Monsieur le Premier ministre, depuis le début de l'épidémie, les sénateurs ont eu la sagesse de ne pas entraver sans motif votre action, mais cette sagesse n'oblige pas au silence. Vous avez fait des soignants des héros nationaux. Vous avez justifié vos décisions par des avis scientifiques. Mais ne soyons pas dupes la parole des médecins a été muselée par la doctrine administrative. Les médecins ont été transformés en agents de l'État et la médecine libérale en médecine officielle. Le 25 mars dernier, vous avez signé un décret qui a tué la liberté de prescrire vous avez imposé des protocoles de soins et vous en avez méprisé d'autres. Pour cela, vous avez invoqué l'absence d'essais cliniques convaincants, face à des médecins de renom. Alors, examinons ce qui est selon vous un essai clinique convaincant : je veux parler de Discovery, lancé le 22 mars dernier. La seule chose que Discovery aura permis de découvrir, c'est l'ampleur d'un fiasco. Alors que 3 200 patients européens étaient

de dissimuler la pénurie d'autres produits. Tout médecin, et j'en suis, sait ce que cela signifie. Monsieur le Premier ministre, vous avez contraint les médecins à violer leur serment d'Hippocrate. Par respect pour les 27 000 victimes de l'épidémie, quand allez-vous rendre aux soignants leur liberté de prescrire et redonner sa dignité à la médecine, en abrogeant le décret du 25 mars ?

Les dernières études qui ont été publiées et validées ne sont pas en faveur de l'utilisation en pratique courante d'un traitement à base de chloroquine en mono-ou bithérapie. Les études se poursuivent néanmoins sur l'ensemble

Ma question s'adresse à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances. Elle porte sur la situation et sur l'avenir de l'industrie pharmaceutique française. La crise du coronavirus a aggravé la pénurie de médicaments en France. Cette situation risque de se dégrader encore à l'avenir. Dans mon département de Lot-et-Garonne, par exemple, l'entreprise UPSA a été en première ligne durant la crise pour accroître la production de Dafalgan et d'Efferalgan. Elle a ainsi assuré la continuité de l'accès des Français au paracétamol. Pourtant, les mesures sanitaires ont entraîné une augmentation des coûts de production. Et comme si cela ne suffisait pas, le prix du paracétamol devrait baisser à partir du 1juin. Dans ces conditions, UPSA continuera-t-elle de produire en France ou va-t-elle se délocaliser, comme tant d'autres l'ont déjà fait ? Cet exemple illustre bien l'absence de vision que nous avons en la matière dans notre pays, et ce depuis de très nombreuses années. La crise du Covid-19 a révélé à quel point nous étions devenus dépendants de l'étranger. Il y a dix ans, il manquait 40 médicaments en France. Aujourd'hui,

Il faut donc en avoir une approche plus stratégique. Madame la secrétaire d'État, concernant UPSA, envisagez-vous une annulation de la baisse du prix du paracétamol ou,, le report de son entrée en vigueur à 2021 ? Plus globalement,

Comme vous le savez, ils ont été fortement mobilisés ces dernières semaines et ont permis de soutenir les efforts de nos soignants, qui étaient en première ligne.

: accélérer l'accès au marché des innovations thérapeutiques, mais également avoir une vision industrielle, notamment dans la politique du médicament. C'est précisément cette vision qui nous a conduits, une première fois, je le signale, à reporter

par la crise du Covid-19. À travers elle, c'est la vitalité de nos territoires qui est en jeu, en particulier du fait de la fermeture de nombreux lieux culturels et de l'annulation des festivals.

Paris. Les mécanismes de l'intermittence demeurent toutefois complexes et la multitude des situations personnelles appelle des mesures précises, circonstanciées et prudentes, prises en concertation avec les acteurs directement concernés. Aussi, monsieur le ministre, deux points majeurs méritent d'être précisés. Le premier concerne la fameuse date anniversaire ouvrant droit au mécanisme d'indemnité de l'intermittence. La prolongation des droits

en effet à craindre que de nombreux projets prévus pour 2020 ne puissent pas être tous réalisés d'ici à l'été 2021. Le second point concerne l'intervention des intermittents au sein du système éducatif. Les heures de l'éducation artistique et culturelle sont globalement plafonnées plafonnées à 70 heures. Si elles sont intégrées dans le calcul des 507 heures minimales exigées, elles restent assujetties au régime général, faisant de fait baisser le calcul global des indemnités des intermittents. Ne conviendrait-il pas, monsieur le ministre, d'augmenter le volume d'heures d'éducation artistique et

Les artistes et les techniciens des secteurs du spectacle, de l'audiovisuel et du cinéma, qui sont les forces vives de la culture dans nos territoires,

du mois d'août 2021, ainsi que, monsieur le sénateur, le report d'autant des dates anniversaires des calculs des droits des intermittents du spectacle. Les modalités

alors que la Commission européenne a autorisé la France à octroyer une aide de 7 milliards d'euros à Air France, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a évoqué la mise en place d'un plan de soutien à l'aéronautique, conditionné par des mesures écologiques et impliquant la suppression de lignes intérieures.

en particulier dans certains territoires fragiles, était subordonnée à l'existence de ces liaisons aériennes. C'est précisément la raison pour laquelle ces lignes, dites « d'aménagement du territoire », bénéficient d'un soutien de l'État et des collectivités territoriales pour combler leur déficit Or les nouvelles normes sanitaires imposées aux compagnies aériennes auront pour conséquence directe un moindre remplissage des avions, ce qui aggravera leur déficit d'exploitation, et une hausse du prix du billet, lequel est déjà très élevé pour les passagers. Les aides financières des collectivités sont déjà extrêmement lourdes pour leurs budgets, alors qu'elles sont elles-mêmes fragilisées par la crise sanitaire. Dans les départements excentrés et difficilement accessibles en train, la relance économique est liée à une reprise rapide rapide de ces liaisons aériennes, attendue par tous les acteurs économiques. Monsieur le secrétaire d'État, l'aide de l'État doit aussi signifier que les avions volent pour remplir une mission de service public.

Nous avons toutefois pris des mesures fortes de soutien aux territoires et aux opérateurs. Tout d'abord, nous avons suspendu les pénalités pour les vols non faits, qui ne sont pas imputables aux transporteurs.

de trésorerie des opérateurs. Enfin, vous évoquez la question importante des contraintes liées aux règles sanitaires dans le secteur aérien. Le décret qui a été publié hier soir prévoit des mesures strictes en termes de protection sanitaire : port du masque obligatoire,

caissières, éboueurs. Le masque est désormais obligatoire dans les transports, à juste titre, pour se protéger et protéger autrui. Alors que, depuis le début de la pandémie, les masques font cruellement défaut, notamment pour les personnels de santé et du secteur médico-social,

Ah ! Aux 100 millions de masques distribués aux soignants et aux malades au travers des circuits organisés par le ministère de la santé, dans les hôpitaux, les Ehpad et les pharmacies,

et aux publics les plus précaires. Ces chiffres ne prennent pas en compte tous les masques délivrés par les collectivités locales. J'ai encore travaillé avec certains d'entre vous la semaine dernière

Pour le reste, les masques sont effectivement largement accessibles dans les petits commerces, les pharmacies, auprès de la grande distribution, comme vous l'avez mentionné. Nous veillons,

volonté politique, mais visiblement, vous ne l'avez pas

Depuis hier, des milliers d'écoliers reprennent progressivement le chemin de l'école tandis que bon nombre d'entre eux restent chez eux. Vous le savez, monsieur le ministre, l'inquiétude est grande parmi les enseignants, les parents, les enfants, mais aussi les décideurs locaux. Bien souvent, les protocoles sanitaires sont difficilement applicables, et ce malgré toute la bonne volonté et le dévouement des personnels municipaux et de l'éducation nationale. Le conseil scientifique lui-même estimait que cette rentrée si particulière était prématurée.

non pas pour des raisons politiciennes, mais en responsabilité, compte tenu des capacités de leurs bâtiments, des effectifs à leur disposition et des protections qu'il est certaines académies ont clairement fait comprendre à ces élus que leur choix entraînerait des conséquences fâcheuses : les enfants des personnels soignants ne seraient plus accueillis dans leurs écoles et aucun enseignant ne serait disponible pour y assurer l'éducation de ces enfants. Voilà de quoi forcer la main aux édiles réfractaires

Depuis le 11 mai, quelques milliers de personnes, principalement des agents de l'assurance maladie, sont investies d'une mission : celle d'enquêter, autour d'un cas positif signalé par le médecin traitant en première ligne, afin d'identifier les chaînes de transmission pour mieux les briser. Ma première question porte sur les garanties que vous pouvez apporter en matière de respect du secret professionnel de la part des professions non médicales- les médecins sont très sensibles sur ce sujet sujet -, et de conservation dans le temps des informations transmises, voire de leur utilisation potentielle à des fins non strictement liées aux soins ou épidémiologiques. En déposant, en décembre dernier, une proposition de loi relative à la sécurité sanitaire, je ne pensais pas que le sujet deviendrait aussi rapidement d'actualité. Je ne pensais pas non plus qu'il prendrait une telle tournure politique, encore que, à bien y réfléchir, on doive s'attendre à des réactions vives dès lors qu'on touche aux libertés individuelles. Ma deuxième question est donc la suivante : ne serait-il pas utile d'inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale afin de sortir d'un régime de l'urgence pour entrer dans un régime de droit commun ? Ne serait-il pas opportun de classer le Covid-19 dans le tableau des maladies à déclaration obligatoire, et de permettre ainsi directement à l'agence régionale de santé (ARS) de déclencher l'enquête autour du cas déclaré ? Enfin, que pensez-vous des prises de position du Conseil constitutionnel sur le fonctionnement des brigades sanitaires et sur la sécurité de nos territoires ultramarins, qui comptaient sur le dispositif de mise en quatorzaine pour protéger la population locale ? La parole

et des libertés (CNIL). Notre unique objectif est de prévenir et de protéger les personnes qui sont ou qui auraient été en contact avec une personne testée positive afin de circonscrire les risques de propagation de l'épidémie et d'éviter le retour à des mesures de confinement strict appliquées à toute une population. Les brigades sanitaires chargées de retracer les contacts des patients infectés par le Covid-19 comportent trois niveaux : le premier est celui du médecin, le deuxième, celui de l'assurance maladie qui dispose de collaborateurs

Du fait de ses relations quotidiennes avec les médecins, l'assurance maladie dispose déjà de beaucoup de données de santé. Les personnels non soignants qui auront accès à ces données sont des collaborateurs dont c'est déjà la mission. Aucune donnée médicale sensible n'a vocation à être partagée au-delà.

Les Républicains. Ma question s'adresse à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice. Madame la garde des sceaux, si l'heure du déconfinement a sonné pour une grande partie de la population active, l'activité du personnel judiciaire ou pénitentiaire ne s'est quant à elle jamais véritablement arrêtée en vertu de la nécessaire continuité de la justice. De la même façon que le personnel soignant, les éboueurs ou encore les caissières, chaleureusement applaudis tous les soirs pour avoir maintenu leur activité au service de la société, les avocats ont ont continué à défendre le justiciable dans le cadre des comparutions immédiates, et souvent malgré le manque de masques et de matériel sanitaire dans les lieux de rétention de liberté. Pourtant- vous le savez, madame la garde des sceaux -près de 40 % des avocats sont susceptibles de quitter leur profession dans les prochaines semaines en raison des graves difficultés de trésorerie occasionnées par leur suspension d'activité. Je veux aussi évoquer la situation des magistrats, qui ont été un maillon important de cette continuité judiciaire. Dans une note du 5 mai, vous avez entièrement laissé aux chefs de juridiction territoriale la responsabilité de décider des mesures de sécurité à respecter, sans pour autant les doter des moyens matériels suffisants. Je souhaite enfin aborder la situation des prisons, en soulignant l'engagement et le professionnalisme de toute l'administration pénitentiaire, notamment des surveillants qui ont dû exercer leur mission dans un contexte sanitaire d'autant plus contraignant. La libération au cours des deux derniers mois de plus de 10 000 détenus, parfois remis en liberté conditionnelle sans avoir pu bénéficier d'une audience dans les délais, pour des raisons liées au Covid-19, suscite des interrogations sur la bonne exécution des peines. peines. Mes questions sont simples, madame la garde des sceaux : avez-vous des solutions solides de soutien à destination des avocats ? Allez-vous enfin imposer le port du masque aux personnels judiciaires et aux justiciables sur l'ensemble du territoire ? Allez-vous organiser un test systématique et massif pour les agents de la pénitentiaire ? Enfin, était-il raisonnable de procéder à la libération d'un tel volume de personnes incarcérées sans garanties solides de réinsertion ?

Enfin, vous évoquez la question des établissements pénitentiaires. Depuis le 28 mars, l'ensemble des surveillants pénitentiaires qui sont en contact étroit

Alors que les Français tentent de reprendre progressivement un rythme de vie ordinaire, les craintes pour notre économie hantent les esprits. Une vieille marotte libérale a refait surface dans les débats ces derniers jours, brandie comme la seule solution à la crise économique qui suivra inévitablement cette crise sanitaire. Cette solution est la remise en cause des 35 heures, responsables, selon certains, de tous les maux dont souffrirait notre compétitivité. Le Gouvernement n'a pas vraiment fermé la porte à cette éventualité. Pourtant, tout au long de cette période, des Français ont travaillé plus, souvent au péril de leur vie. Nous ne pouvons demander aux caissiers, aux éboueurs, aux soignants, aux routiers, à toutes celles et tous ceux qui ont été les premiers de tranchée, de payer doublement l'effort de guerre en leur enjoignant d'allonger leur temps de travail. Quelle drôle de manière de leur témoigner notre reconnaissance que de leur proposer un monde d'après plus injuste et plus rude encore que celui d'avant Aujourd'hui, de nombreux citoyens sont au chômage partiel, ont ou vont perdre leur emploi. La priorité de ce gouvernement doit être d'empêcher le chômage de masse et le risque de centaines de milliers de sans-emploi supplémentaires. La question obsédante n'est donc pas celle du « travailler plus » individuellement, mais celle du « travailler tous ». Aussi, madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer très clairement si le Gouvernement a, oui ou non, le projet de remettre en cause les 35 heures ? de privilégier le retour à l'emploi de tous les Français par la concertation et le dialogue social ?

Faute d'action forte en faveur de l'apprentissage, de nombreux métiers manqueront de main-d'oeuvre qualifiée dans les prochaines années. Un premier constat établi pendant le confinement fait état d'une baisse potentielle des candidats à l'apprentissage autour de 30 %. Portes ouvertes annulées, rencontres physiques impossibles : des élèves s'orientent vers les filières générales, quand ils n'y sont pas contraints en raison de la défection des maîtres de stage. En effet, des entreprises, fragilisées par l'arrêt brutal de leur activité, renoncent aujourd'hui à recruter des apprentis. Avec la baisse du nombre d'apprentis, des centres de formation vont être confrontés à des problèmes de financement, puisque celui-ci dépend du nombre d'apprentis. Avec la baisse du nombre d'apprentis, des centres de formation vont être amenés à fermer des classes, des spécialités et des niveaux d'études et à réduire le nombre de formateurs. À terme, cela se traduira par un déficit de compétences pour des métiers qui déjà peuvent se trouver en tension actuellement. actuellement. Madame la ministre, je vous soumets donc deux questions relatives à l'apprentissage, voie de la réussite. La première est portée par mon collègue Olivier Henno : quels outils comptez-vous mettre en place pour accompagner les entreprises qui font le choix de recruter et de maintenir des apprentis ? Par pouvez-vous envisager dès aujourd'hui pour la rentrée prochaine et pour une durée limitée d'élargir le statut de scolaire alternant aux candidats à l'apprentissage qui ne parviendraient pas à trouver une entreprise ? La parole

Merci